Parents, élèves et enseignants ont découvert en janvier dernier une carte scolaire actant sans concertation 1 000 suppressions de postes en primaire et 500 dans le secondaire. Les mobilisations se multiplient un peu partout.

337 postes et 240 classes supprimées ! Cela fait suite, qui plus est, au scandale de la fermeture de sept lycées professionnels parisiens, décidée par Valérie Pécresse avec l'aval de votre ministère. Le problème n'est pas limité à la capitale. Les banlieues comme les zones rurales sont durement frappées. Entendez-vous l'appel des maires ruraux, lesquels demandent un moratoire immédiat sur les fermetures de classes et d'écoles ? Monsieur le ministre, pendant la crise de la covid-19, le Gouvernement nous expliquait que le temps éducatif devait être protégé comme la prunelle de nos yeux ... Aujourd'hui, vous jetez cela aux oubliettes. L'éducation nationale redevient une cible prioritaire des coupes budgétaires.

l'occasion de dire dans cet hémicycle que nous allons perdre environ 500 000 élèves dans les cinq années à venir. La situation est plus aiguë encore à Paris, puisque la baisse de la natalité se combine

Nos critères pour assurer la répartition des postes sur le territoire sont simples : équité et universalité. Ma responsabilité est bien celle de l'équité territoriale et celle-ci amène à faire des choix, des choix, pour que le service public d'éducation soit préservé sur le territoire français et pour que nos professeurs soient mieux rémunérés. En effet, la hausse du budget de l'éducation nationale est de 6,5 % cette année ; pour mémoire, elle était de 2 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2017.

Certains usagers posent même la question de notre capacité à accueillir cet événement ! Cette semaine, vous avez visité le chantier Éole, grand projet de prolongement du RER E vers l'ouest parisien. Je me félicite que l'État puisse accompagner la région d'Île-de-France pour de tels

Dès 2024, c'est-à-dire demain, 600 millions d'euros manqueront à l'appel pour financer le fonctionnement des nouvelles lignes actuellement en chantier. Le réseau francilien va en effet doubler d'ici à 2030, pour des besoins en financement Il y a trois ans, la chambre régionale des comptes tirait déjà la sonnette d'alarme au sujet de la gestion inadaptée et déséquilibrée d'Île-de-France Mobilités. L'endettement de cet opérateur, après avoir été multiplié par sept entre 2013 et 2018, a encore augmenté de 64 % pour la seule année 2022. face aux difficultés accumulées, l'État est de nouveau venu au secours d'Île-de-France Mobilités, en abondant son budget de 200 millions d'euros. Malgré cela, Île-de-France Mobilités a décidé d'augmenter le prix du passe Navigo pour un service qui continue de se dégrader, notamment pour les RER B

d'accueillir correctement des millions de visiteurs et de permettre aux Franciliens qui travaillent d'avoir des transports à l'heure, suffisants et de qualité ? La parole

Courageusement, les députés de la majorité gouvernementale ont quitté l'hémicycle au moment du vote sur ce texte, ce qui en dit long sur leur respect de la démocratie parlementaire ... Plus profondément encore, madame la Première ministre, cette attitude est le reflet de l'impensé politique du Gouvernement s'agissant de son projet industriel pour EDF comme de ses objectifs concrets de réforme du marché de l'électricité dans l'intérêt général des Français et de toutes nos entreprises. Madame la Première ministre, si ce texte, à présent déposé sur le bureau du Sénat, ne vous convient pas, quelles sont vos propositions de substitution pour EDF ? Comment entendez-vous répondre immédiatement aux difficultés de nombreuses d'entreprises dont l'existence est en jeu

Je ne vois pas ce qu'il apporte, parce que nous avons engagé la prise de participation d'EDF par l'État à hauteur de 100 % ; au moment où je vous parle, nous détenons

d'argent public du contribuable soient mis à contribution pour les soutenir face à la crise de l'électricité ? Je pense que c'est tout simplement un gigantesque gaspillage d'argent public

ne se profile en France et en Europe. Ce qui est ici en question, c'est la capacité du Président de la République et de votre gouvernement à peser sur la réforme du marché de l'électricité dans l'Union européenne. L'entreprise nationale EDF doit être au coeur de la reconquête de la souveraineté économique française.

Parce que cela ne relève pas de votre délégation, je ne vous interrogerai pas sur l'augmentation de la cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), que vous souhaitez imposer aux employeurs territoriaux à compter de 2024 et à laquelle ils s'opposent fermement. En revanche, parmi les sujets qui semblent des angles morts de votre réforme, il y a les effets que peut avoir le recul proposé de l'âge légal de départ à la retraite sur l'engagement politique et associatif local. En effet, la retraite est l'occasion pour bon nombre de personnes de franchir le pas d'une candidature à l'élection municipale de leur village ou d'être administrateur et bénévole d'une association culturelle, sportive ou sociale.

Du côté de l'engagement politique, à la suite des élections municipales de 2020, le nombre de maires de plus de 60 ans a atteint 55 %. En somme, être retraité, c'est endosser un rôle non négligeable dans la cohésion sociale de notre pays, qui plus est lorsque l'on sait que ce sont les profils les plus assidus dans leurs missions bénévoles et fonctions électives, du fait de leur disponibilité. Malgré tout, nous devons considérer que cette situation est fragile, car les difficultés de renouvellement des équipes sont déjà perceptibles, en raison d'un statut de l'élu local et de droits des bénévoles inadaptés à notre époque. Aussi, avez-vous anticipé et évalué les conséquences de votre réforme sur la dynamique de l'engagement ? La parole

de votre question. Vous m'interrogez sur la prise en compte du bénévolat dans la réforme des retraites. Il est vrai que l'engagement associatif constitue l'une des pierres angulaires de la cohésion de notre société. L'engagement bénévole, notamment pour les responsables d'associations, exige du temps et de l'énergie. Alors, oui, réfléchissons à la manière de valoriser et d'encourager

plus, le financement de trimestres de retraite peut rapidement devenir une charge difficile à assumer pour les associations qui sont concernées. Plus généralement, il nous appartient de veiller au caractère contributif et à l'équilibre de notre système de retraite. C'est la raison pour laquelle les modalités d'acquisition de droits à la retraite pour les bénévoles doivent faire l'objet d'une analyse approfondie, pour en assurer la bonne mise en oeuvre. Nous espérons que les débats en cours à l'Assemblée nationale permettront d'aborder ce sujet au travers des différents amendements qui sont déposés à l'article 7. Je pense en particulier à un amendement du groupe Renaissance, qui vise à évaluer l'opportunité d'accorder des droits supplémentaires à la retraite aux responsables associatifs. Par ailleurs, sans avoir posé de question à ce sujet, vous avez abordé le

contribueront légèrement davantage, leur taux de cotisation passant de 30,65 % à 31,65 % l'année suivante. Cette hausse d'un point reste largement inférieure au taux de cotisation implicite dans la fonction publique d'État, qui est de l'ordre de 74 %.

Lundi dernier, nouveau fait du prince, les salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont appris le démantèlement de leur institution, pourtant reconnue internationalement. La surprise fut totale, créant sidération et inquiétude chez ces 1 700 salariés.

C'est un garde-fou institutionnel mis en place après la catastrophe de Tchernobyl et dont l'utilité a été prouvée après Fukushima. Alors que vous relancez un programme nucléaire d'ampleur, il nous paraît essentiel de ne pas casser une organisation qui a fait la preuve de son efficacité. Pourquoi voulez-vous démanteler l'IRSN ? Est-ce une demande de l'exploitant, dès lors que les exigences de sûreté réclamées par l'Institut, qui ne répondent, je le rappelle, qu'aux seules considérations scientifiques, lui paraissent trop élevées ?

Pourquoi écarter la représentation nationale de ces choix essentiels ? Pour accélérer le nucléaire, vous n'avez pas à affaiblir les exigences de sûreté. La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur

De tels blocages causent de graves préjudices. Un parcours du combattant commence pour les usagers, qui, dans une pagaille monstre, doivent trouver des solutions de substitution pour répondre à l'urgence et se faire rembourser leur billet.

12 milliards d'euros ont été perdus à cause de ces blocages ; la France était à l'origine de 97 % des perturbations aériennes au sein de l'Union européenne.

Il convient d'assurer la continuité du service public en soumettant le droit de grève des contrôleurs aériens à un système de notification préalable de 48 heures, comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les autres professions du monde aérien.

! Madame la ministre, remplissez pleinement vos fonctions, personne ne vous en empêche, et laissez l'Arcom faire son travail

330 000 personnes sans logement sur notre territoire, des milliers d'adultes et d'enfants refusés chaque soir par le 115 pour un hébergement d'urgence, près de 4 millions de Français mal logés ... Cette situation est indigne dans notre pays, où, force est de le constater, les fractures ne cessent de s'aggraver. Sont en cause des évolutions conjoncturelles : la crise sanitaire avait déjà fragilisé les plus précaires, l'inflation les a ensuite atteints de plein fouet. Aujourd'hui, les dépenses énergétiques deviennent insoutenables insoutenables pour de nombreux ménages modestes. La situation s'explique également par des raisons structurelles. Les prix à l'achat et à la location n'ont cessé de grimper depuis trente ans. Et l'effort public pour le logement en France n'a cessé de chuter depuis 2010. On le sait, le logement est le premier sujet de préoccupation des Français. Il devient également une source aggravante d'exclusions et d'inégalités. À titre d'exemple, j'évoquerai la situation des mères de famille monoparentale 40 % des femmes avec un enfant vivent dans de mauvaises conditions de logement, contre 20 % pour la moyenne de la population. Vous allez probablement me dire, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas responsable de l'état du mal-logement en France, qui perdure depuis trop d'années, mais vous êtes aujourd'hui responsable du changement de braquet, du tournant à prendre pour permettre à tous les Français de se loger dignement. Monsieur le ministre, allez-vous enfin relancer la construction de logements neufs, particulièrement de logements sociaux ? Allez-vous renouer avec l'objectif de 500 000 logements neufs par an ? La parole

République dès 2017. Il a permis à plus de 450 000 personnes de sortir de la rue et d'avoir un toit. Dans le même temps, la situation sociale, économique

plusieurs économistes commencent à s'inquiéter de l'affaire. Et ils ont raison ! Ainsi, Rexecode nous dit que, de 2019 à 2022, la France a perdu des parts de marché et dégradé son solde extérieur dans presque tous les secteurs industriels.

enregistré un excédent record de plus de 50 milliards d'euros, tout comme la balance des revenus, avec un excédent de plus de 31 milliards d'euros. Le déficit commercial, ce n'est pas que la balance des biens, c'est également la balance des services et la balance des revenus. Ainsi, les chiffres sont évidemment bien moindres que ceux que vous annoncez sur le déficit commercial. Ils sont de l'ordre de 50 milliards d'euros. Comment comptons-nous agir pour réduire le déficit de la balance des biens ?

fut une grande réussite. Elle a permis à de nombreux Français de dire pacifiquement, sereinement et avec détermination leur opposition résolue à ce texte. Cette mobilisation a d'ailleurs été très forte dans les villes moyennes,

Les Français ont compris votre opération d'illusionniste : il n'y aura pas de pensions à 1 200 euros, sauf pour une très faible minorité. Duperie également pour ce qui concerne la situation des femmes, qui sont les principales victimes de votre réforme, tout comme les catégories populaires ayant commencé à travailler tôt. Votre gouvernement est décidément toujours doux avec les puissants et dur avec les plus fragiles ! Le Président de la République, le Gouvernement et sa majorité de circonstance sont, hélas ! totalement sourds au mouvement social sans précédent qui traverse notre pays. Face aux syndicats, le Gouvernement a agité le spectre des blocages à la veille des vacances, pour tenter de retourner l'opinion. Pourtant, ce sont bel et bien le Président de la République, le Gouvernement et sa majorité qui bloquent le pays. Quelles seraient les conséquences si votre néfaste projet suivait son cours, sans tenir compte de son rejet très majoritaire dans le pays ? Quand allez-vous prendre la seule et unique décision susceptible d'apaiser le pays, à savoir le retrait de votre projet de réforme et l'ouverture de véritables négociations avec les partenaires sociaux ?

de votre camp face à une réforme qui vise à équilibrer dans la durée un système par répartition en demandant un effort aux Français une augmentation progressive de la durée de travail tout au long de la carrière. Madame la sénatrice,

en fonction de la durée de cotisation et du niveau de revenu tout au long de la carrière, comme la Première ministre l'avait annoncé lors de sa conférence de presse inaugurale. C'est faux ! Hier, l'Assemblée nationale, légitime dans son exercice, a décidé de rejeter l'article 2 du projet de loi.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain restera très mobilisé contre cette réforme, avec responsabilité et dans le respect du débat. Mesdames, messieurs les ministres, écoutez les Français et écoutez les élus.

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et a trait à la remise en cause des chantiers de renaturation des cours d'eau. Le décret du 30 juin 2020 a très largement simplifié les procédures préalables à l'engagement de ce type de travaux, en soumettant ceux-ci non plus à autorisation, mais à déclaration. des milieux aquatiques et prévention des inondations) de mettre en oeuvre de nombreux chantiers de renaturation des cours d'eau, en redonnant un fonctionnement naturel aux cours d'eau, en restaurant les continuités écologiques, en améliorant la richesse et la variété des espèces et des habitats, en renforçant la capacité de rétention des crues et la réduction des inondations. Or un arrêt du Conseil d'État du 31 octobre 2022 a annulé l'article du décret du 30 juin 2020 qui simplifiait grandement les procédures préalables aux travaux de renaturation. Aujourd'hui, les présidents de syndicat mixte, s'ils ne demandent pas le rétablissement à l'identique du texte invalidé par le Conseil d'État, souhaitent que les opérations de renaturation n'aggravant pas le risque d'inondation, n'affectant pas les moulins, ne présentant pas de danger pour la sécurité publique

plébiscités par les élus, les populations et les associations de défense de l'environnement. En l'état, le maintien d'un tel arrêt et la suppression du « système déclaratif » feront de 2023 une année blanche en matière de travaux de renaturation, alors même que leur financement est assuré et que de nombreuses entreprises de travaux publics attendent le lancement de ces opérations. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous faire pour que le bon sens l'emporte ? La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le le sénateur Hugonet, je vais faire très exactement ce que vous me suggérez. Le Gouvernement va prendre un nouveau décret,

Voilà dix jours, j'étais au coeur du Donbass, où j'ai eu le privilège d'avoir un contact direct avec des combattants ukrainiens revenant du front ou, plutôt, des tranchées. c'est Verdun au XXI siècle : froid, boue, puanteur, rats, tirs d'artillerie continus et vagues répétées de chair à canon russe, qu'il faut sans cesse contenir puis repousser. de ces combattants, dont la seule préoccupation est de survivre. Pour cela, ils ont plus que jamais et urgemment besoin de nous, de notre technologie, de nos armes, dont le canon Caesar que nous avons vu en action et qu'ils louent pour son allonge, sa précision et sa mobilité. Allons-nous enfin accélérer la cadence de livraison des obus et des pièces détachées, qui leur font si terriblement défaut, ainsi que des douze Caesar supplémentaires prévus ? Allons-nous livrer les blindés légers AMX 10 RC promis ? Si oui, quand et combien ?

Monsieur le sénateur, je connais votre engagement sur ces sujets et vous suis reconnaissante de les évoquer devant nous aujourd'hui. Dans le cadre du soutien que la France octroie à l'Ukraine, nous examinons trois critères fondamentaux à chaque fois que nous procédons à une cession d'armes à ce pays. apportée aux priorités des demandes des Ukrainiens, dans une logique défensive et dans la maîtrise du risque d'escalade. Le deuxième est la préservation de notre modèle de sécurité et de défense. est l'efficacité opérationnelle rapide des capacités fournies, avec des équipements fonctionnels, une formation adaptée, des munitions et le MCO (maintien en condition opérationnelle). Nous répondons rapidement aux priorités des demandes ukrainiennes sur les blindés de combat, l'artillerie et la défense sol-air. Les canons Caesar sont une réponse adaptée. Dix-huit canons sont déjà livrés et seront complétés rapidement par de nouveaux canons français et danois. La France a par ailleurs donné des LRU, avec des lots de roquettes. De même, pour la défense sol-air, nous avons déjà livré des missiles Mistral et des batteries Crotale. Nous poursuivrons l'aide à la protection du territoire ukrainien

AMX 10 RC, qui iront bientôt en Ukraine. Par ailleurs, nous avons créé avec le Parlement un fonds spécial de soutien de 200 millions d'euros, qui sont déjà bien utilisés. Ce fonds permet à l'Ukraine

Saint-Martin-Valmeroux, Ydes, les Ternes, Murat, Saint-Flour, sont les victimes de l'année. Avec cette même logique inacceptable, beaucoup d'autres suivront ! Cette année, nous sommes en plus victimes d'un marché de dupes, qui consiste à accroître les moyens de votre ministère de 6,5 %, malgré la baisse des effectifs, et de constater les réductions de moyens sur nos territoires ! Tout cela sans concertation, sans délai de prévenance, avec une méthodologie remontant à la III République, sans laisser le temps aux familles et aux élus de s'organiser, en ignorant les initiatives prises sur les territoires et les investissements réalisés par les maires. Monsieur le ministre, si vous voulez vraiment réduire nos moyens, bien qu'on augmente les vôtres, ne le faites pas au détriment des élèves et des effectifs présents devant ces élèves. dans le Cantal, seulement 670 enseignants du premier degré sur 780 sont devant des élèves, soit un ratio de 85 %, sans parler des effectifs administratifs. Monsieur le ministre, avez-vous l'intention d'améliorer ce ratio, en remettant des enseignants devant nos élèves des classes rurales, pour ne pas envoyer un signal mortifère à nos petites écoles, qui sont la vie de nos communes ? La parole

la France est confrontée à un problème de natalité qui n'épargne pas, malheureusement, votre département. Cette situation nous amène en effet à procéder à des ajustements dans la carte scolaire, selon deux principes, un principe d'équité territoriale - nous accompagnons les territoires qui gagnent des élèves, en créant des postes de façon substantielle

Nous tenons donc nos engagements, y compris celui du Président de la République de ne fermer aucune école en milieu rural sans l'accord du maire. Par ailleurs, c'est l'objet de l'augmentation du budget de l'éducation nationale que vous avez mentionnée, nous avons prévu d'accroître la rémunération des professeurs

la préparation de la carte scolaire 2023-2024 se traduit par des suppressions importantes de postes, particulièrement dans le premier degré, comme cela vient d'être Dans de nombreux départements, la rentrée sera donc, une fois de plus, compliquée. En Haute-Vienne par exemple, de nombreuses fermetures de classes et suppressions de postes sont prévues alors même que le taux d'encadrement y est inférieur à la moyenne nationale. La baisse du nombre d'élèves accueillis ne saurait tout justifier. L'élaboration de la carte scolaire ne peut être dictée par de simples considérations comptables. Monsieur le ministre, l'école publique est en bien mauvais état. Le constat est cruel, mais, hélas ! sans appel sur tous les territoires, ruraux comme urbains, en région comme à Paris, dans le primaire comme dans le secondaire des classes, sans enseignants pendant plusieurs jours, transformées en garderie ; des brigades de remplacement dont les effectifs sont affectés à d'autres missions ; des enfants en situation de handicap accueillis sans moyens supplémentaires, c'est-à-dire sans véritable possibilité d'inclusion. Un tel état des lieux justifierait, à lui seul, un moratoire sur la fermeture de classes. Au-delà se pose la question des moyens que nous voulons donner à l'école publique pour assurer l'avenir de nos enfants. Monsieur le ministre, comptez-vous sortir de la logique comptable afin de doter l'éducation nationale des moyens indispensables aux besoins des enfants, des enseignants et des territoires ? La parole

je ne reviendrai pas sur la question démographique, sauf pour noter que, dans votre département, la baisse du nombre d'élèves sera de 400 enfants à la rentrée. Je vous rappelle, en outre, que la préparation des mesures de rentrée est un travail qui commence très en amont. Il comporte plusieurs phases d'échange et de dialogue avant que des décisions définitives ne soient prises au mois de juin et au mois d'août. À l'heure actuelle, les décisions définitives ne sont donc pas encore prises. (Dasen), les recteurs, les inspecteurs d'académie, nous sommes encore dans cette phase de dialogue et d'échange. Nous fermons des classes, c'est vrai, mais nous en ouvrons aussi beaucoup. Je suis convaincu, comme vous, que l'école est un facteur de dynamisation des territoires. Ce travail doit être mené, je vous l'accorde, entre les élus locaux et l'éducation nationale. Dans dix académies, nous avons créé les territoires éducatifs ruraux, qui permettent d'unir les forces de l'éducation nationale

Enfin, madame la sénatrice, je me permets de vous faire remarquer à propos des moyens de l'école que la hausse de 6,5 % du budget, soit 3,7 milliards d'euros, constitue une augmentation considérable, qui nous permettra de mieux payer les professeurs et, par conséquent, de pourvoir les postes

Monsieur le ministre, la fin de votre réponse est un peu facile, mais les faits sont là ! Promouvoir l'égalité des chances, lutter contre les fractures territoriales, émanciper et former de futurs citoyens, telles sont les missions de notre système éducatif. Monsieur le ministre, notre école va mal, la méthode doit changer. Vous l'avez d'ailleurs souligné, tout est question de choix : ce n'est pas en supprimant des postes que notre école publique ira mieux

naître ou ne plus naître à Autun, telle est désormais la question qui angoisse les 62 000 habitants du Morvan, entre Saône-et-Loire, Nièvre et Côte-d'Or, après votre annonce de la fermeture de la maternité d'Autun. Cette fermeture provoque un vent de colère et de révolte chez les équipes de soignants, ô combien dévoués, mais aussi chez les élus locaux et la population, devant ce qui est vécu comme un nouveau « déménagement » du territoire. Cette fermeture suscite l'inquiétude des femmes enceintes, désormais contraintes de parcourir plus d'une heure, voire une heure trente de route, pour se rapprocher d'une maternité, alors même qu'une étude réalisée dans notre région a montré combien l'augmentation de cette distance retentissait sur la santé périnatale. Cette fermeture locale doit préoccuper à l'échelon national. Monsieur le ministre, vous avez commencé par la justifier ainsi : « Nous n'arrivons plus à trouver des professionnels pour assurer la sécurité. » Est-ce donc là votre seule politique ? Après avoir fermé une maternité sur trois en vingt ans, votre ministère va-t-il amplifier cette concentration et fermer toutes les maternités de niveau 1 du pays ? Face au tollé provoqué par votre annonce, vous avez renié le mot de « fermeture » dans un tweet qui disait Inexact : les accouchements sont suspendus aujourd'hui par manque de personnel. » Finalement, monsieur le ministre de la santé, est-ce là votre seule ambition face aux pénuries médicales que de demander aux femmes de « suspendre les accouchements » et aux malades de suspendre leur maladie ?

Quelle est la situation actuelle ? Les accouchements sont suspendus à la maternité d'Autun depuis mi-décembre, faute de personnel médical. J'imagine que, comme moi, vous refusez de mettre en danger la santé des parturientes et des enfants parce qu'il n'y aurait pas de personnel compétent pour les prendre en charge.

répondant aux besoins de santé de la population. Il est hors de question, bien entendu, que les femmes du Morvan n'aient pas de solution satisfaisante au moment de leur grossesse. Dans le même temps, nous continuons de travailler avec les élus, les professionnels et les représentants des patients. Plusieurs

Ensuite, nous mettons en place un service de périmaternité à Autun permettant la prise en charge des femmes jusqu'à l'accouchement et tout de suite après l'accouchement, avec une antenne à Château-Chinon pour mieux couvrir l'ensemble du Morvan.

je suis de très près, car il est emblématique de la construction d'une réponse à l'échelle du territoire et non plus simplement de façon focalisée. La parole

Monsieur le ministre, le 1 juillet 2007, la France ouvrait son marché de l'électricité et du gaz à la concurrence pour les particuliers, faisant naître par la même occasion des promesses sur une baisse des prix ainsi que sur un système plus performant et plus lisible pour les consommateurs. ans après, je crois pouvoir dire, au nom de millions de Français, que le poids de l'énergie sur le budget des ménages est aujourd'hui extrêmement préoccupant. Sans surprise, différentes études montrent que le prix de l'électricité a progressé de près de 50 % en dix ans, et ce n'est malheureusement pas terminé ! Même constat alarmant pour le gaz Au final, comme souvent, c'est le consommateur qui fait les frais de la situation actuelle dont les causes sont multiples : guerre en Ukraine, marché européen de l'énergie en difficulté et stratégie énergétique des différents gouvernements souvent incohérente. d'ici au 30 juin 2023, les tarifs réglementés du gaz sont voués à disparaître, obligeant des millions de ménages à renégocier leurs contrats, avec des tarifs qui vont bondir. Alors que la reprise économique s'amorce en Chine et que ce pays va fortement augmenter sa consommation de gaz, il y a fort à craindre que le prix de cette énergie ne s'envole et que le marché mondial ne s'affole. Dans ce contexte, il est urgent de prolonger ces tarifs réglementés pour ne pas plonger des millions de Français dans la précarité énergétique. Monsieur le ministre, ma question est simple : sans créer un nouveau « chèque allez-vous reporter la fin des tarifs réglementés du gaz prévue le 30 juin 2023, sachant que, depuis octobre 2021, la Commission européenne autorise les États à prendre des mesures exceptionnelles pour la protection des consommateurs ? La parole

deux ans, la France, plus qu'aucun autre État européen, protège le consommateur français contre la flambée des prix du gaz et des prix de l'électricité. C'est un échec ! Cela s'appelle le bouclier tarifaire.

Je rappelle, par ailleurs, que sur 12 millions de consommateurs de gaz, 10 millions ont déjà fait le choix de sortir des TRV. Je sais bien que les mots entretiennent la confusion, mais en ce qui concerne l'électricité nous sommes producteurs,

fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Ce prix de référence sera maintenu, quoi qu'il arrive sur les prix du gaz au-delà de juin 2023. Je le redis : la protection tarifaire sera garantie par le bouclier que nous avons mis en place. Monsieur le ministre, dans un environnement de plus en plus dérégulé, le tarif réglementé de vente du gaz reste une référence claire sur le marché. Si le tarif réglementé disparaît, il manquera une balise à laquelle se référer en cette période trouble. La

c'est à s'y méprendre ! Madame le ministre, le 9 février dernier, vous avez clairement menacé de ne pas renouveler les fréquences de chaînes d'information privées depuis les studios d'un média public. Ces propos choquants représentent une atteinte à l'indépendance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle atteinte au pluralisme porté, notamment, par le travail des équipes de C8 et CNews, chaînes suivies quotidiennement par plus de 11 millions de téléspectateurs. Ils sont enfin une menace pour la liberté d'expression et le débat démocratique. Madame le ministre, si vos propos portent les valeurs de la République, ce sont celles d'une République soviétique ou d'une République bananière Dois-je vous rappeler que nous sommes à Paris, pas à Pyongyang ni à La Havane ? Votre atteinte à la liberté d'expression et au débat démocratique est aggravée par un « deux poids, deux mesures » : samedi encore, la chaîne publique France 2, incapable d'égard pour les élus d'opposition, accueillait en vedette un tueur en série, sans réaction de l'Arcom ni de votre part ! Vous avez une conception et une application très sélective du rappel du cadre de la loi ... La chaîne C8 collectionne, elle, près de 6,7 millions d'euros d'amende depuis six ans pour, disons-le,

La vérité, c'est qu'en 2025 nous serons à deux ans de l'élection présidentielle et que vous ne supportez plus que l'opposition puisse s'exprimer sur une chaîne qui, pourtant, fait preuve, elle, d'une véritable pluralité en invitant toutes les opinions

L'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'État sur l'équilibre financier des collectivités locales. » En application de l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation

sénateurs, l'équilibre des relations commerciales au sein de la chaîne agroalimentaire et, à travers lui, la juste rémunération de chacun des maillons de la chaîne, au premier rang desquels nos agriculteurs : tel est le débat auquel nous invite collectivement cette proposition de loi, un débat que vous avez souhaité avoir aujourd'hui, en vous en saisissant pleinement. Ce sujet est d'une actualité forte pour plusieurs filières et plusieurs maillons de notre chaîne alimentaire. Notre défi commun, celui du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, comme du Sénat, j'en suis persuadé, est d'assurer notre souveraineté alimentaire, avec nos agriculteurs et au service de notre pays, de nos concitoyens. Il est aussi de notre devoir collectif- Gouvernement, parlementaires, agriculteurs, industriels, distributeurs, citoyens -, de trouver et proposer des solutions pour nous assurer que nous conserverons une capacité à produire dans tous nos territoires, dans tous vos territoires, pour nous alimenter en qualité et en quantité suffisante dans les décennies à venir. C'est un objectif fondamental qui doit être très largement partagé, car, comme j'ai l'habitude de le rappeler, chacun de ces maillons s'inscrit dans une relation d'interdépendance forte, qui les oblige, ou devrait les obliger, à une responsabilité réciproque. De la capacité de nos agriculteurs à dégager des revenus, ce qui est en soi un enjeu primordial, dépendent aussi la résilience de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire

Je veux revenir sur ces sujets, parce que trop de propos versent trop facilement dans la caricature, souvent dans des enceintes extérieures au Parlement. Ce texte vise à établir un meilleur équilibre des relations commerciales, mais il ne s'agit pas de monter les distributeurs contre les industriels, ou l'inverse. Notre souveraineté alimentaire et la sécurité de nos approvisionnements sont des préoccupations partagées par tous les Français et, il faut le dire, par l'ensemble des maillons de notre chaîne alimentaire. plus vrai dans le contexte que nous connaissons, qui rappelle à chacun, s'il en était besoin, le caractère stratégique de ces objectifs. Notre sécurité et notre souveraineté alimentaires dépendent en fait de chacun des trois maillons de la chaîne, pris individuellement et collectivement. Cette délicate recherche de l'équilibre doit nous inviter tous à la mesure et à la tempérance. Avant d'en venir au texte soumis à votre chambre, je veux rapidement rappeler le chemin qui a été parcouru lors du quinquennat précédent pour améliorer le revenu de nos agriculteurs, rééquilibrer les relations commerciales

À l'aval, le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions en valeur et en volume ont mis fin aux promotions agressives, destructrices de valeur et déroutantes, tant pour les consommateurs que pour les agriculteurs. La loi Égalim 2 est venue renforcer la construction en « marche avant » du prix, si vous me permettez cette expression, depuis le producteur jusqu'au distributeur. À l'amont agricole, le principe est désormais celui d'une contractualisation écrite, pluriannuelle et obligatoire. Concrètement, les contrats doivent comprendre un certain nombre de clauses qui sécurisent les agriculteurs et leur donnent de la visibilité sur leur rémunération. Je pense notamment aux clauses de révision automatique des prix. À l'aval, de nombreuses mesures ont été introduites, comme la transparence et la non-négociabilité de la matière première agricole. Le rééquilibrage des relations a été constaté dès la fin du cycle des négociations commerciales annuelles, qui s'est achevé le 1 mars 2022. Il a bénéficié à nos agriculteurs et à nos transformateurs, en permettant pour la première fois de mettre fin à ce qui avait été constaté par tous depuis dix ans, à savoir la spirale destructrice de la guerre des prix sur les produits agricoles. En particulier, la transparence et la non-négociabilité de la matière première agricole ont donné des résultats très encourageants. Naturellement, Naturellement, soyons modestes, du chemin reste à parcourir et je sais les difficultés qui subsistent, mais les lois Égalim ont contribué au maintien dans nos territoires de nombreuses exploitations agricoles et ont posé clairement la question de la rémunération Les décrets d'application portant sur les relations commerciales sont quasiment tous adoptés, ceux qui étaient indispensables au bon fonctionnement de la loi l'ayant été dès la fin de 2021. Il revient évidemment aux acteurs de s'en saisir pleinement dans un contexte particulier, la guerre en Ukraine étant venue perturber le cycle de négociations. Nous devons donc absolument éviter de fragiliser cet édifice Égalim, dont la mise en oeuvre pleine et entière ne débute que cette année. C'est notamment le cas pour de nombreuses PME qui avaient conclu leurs négociations en 2021, avant l'entrée en vigueur de la loi Égalim 2.

et que ce dispositif expérimental y a, de toute évidence, largement contribué. Suspendre pendant deux ans cette expérimentation serait revenu à l'enterrer. Cette proposition portait donc en elle le risque de relancer la guerre des prix et la destruction de la valeur. sénateurs- c'est une conviction que j'aimerais vous faire partager -, qu'il serait sans doute mortifère de glisser doucement vers un débat qui opposerait revenu des agriculteurs et protection du pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus modestes, comme si l'un ne pouvait s'améliorer qu'au détriment de l'autre.

Au demeurant, et malgré certaines critiques, des enseignements sont quand même à tirer des deux rapports d'évaluation remis au Parlement, qui démontrent que l'effet inflationniste attribuable à ces mesures a été plus que marginal. Je suis persuadé que les dispositifs de contrôle et d'évaluation seront de nature à nous éclairer encore sur ce dispositif SRP+10. Telle est, sans doute, la logique que nous devons privilégier mieux évaluer, avec le Parlement, plutôt que suspendre ce dispositif et prendre le risque d'affaiblir la portée des lois Égalim. Je crois, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, que vous avez su être à l'écoute des inquiétudes qui ont pu être exprimées. Je salue les premières évolutions que vous avez proposées. L'amendement que vous défendrez

ainsi élargir ce dispositif, pourtant conçu pour répondre aux spécificités de la chaîne agroalimentaire, à des produits de consommation et à des acteurs économiques en tout point différents. C'est l'occasion pour moi de rappeler avec force que produire pour nourrir n'est pas une activité comme une autre. Cette singularité, c'est un élément de fierté pour nos agriculteurs, mais aussi pour nous, qui avons conscience que l'agriculture est une part de notre histoire, qu'elle participe à la place de la France dans le monde, à la vitalité et au dynamisme économique des territoires.

Il est donc important pour moi de revenir à l'essentiel : donnons-nous trois années supplémentaires pour évaluer correctement l'expérimentation, prolongée à périmètre constant, en lien étroit avec le Parlement.

et des sanctions alourdies. Nous nous approchons par ailleurs d'un plus juste équilibre, cher à mon collègue ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur l'article 3, qui vise à mieux encadrer les cas où un accord n'a pu être conclu entre distributeurs et fournisseurs au 1 mars. Je tiens à cet égard à souligner le travail extrêmement précis et pointu réalisé par la rapporteure et votre par la rapporteure et votre commission. Plus globalement, je veux saluer la qualité des travaux menés par Mme la rapporteure et Mme la présidente de la commission. Je les remercie des améliorations qu'elles ont contribué à apporter au texte. Elles témoignent de leur engagement et de leur vigilance, depuis longtemps, sur ces questions.

Avant de vous présenter les travaux de la commission des affaires économiques, je tiens à rappeler que c'est tout de même la troisième fois en cinq ans que le législateur est amené à intervenir pour clarifier et renforcer le cadre applicable aux négociations et aux relations commerciales. Pourquoi ? ? Parce que le niveau de tension et de défiance entre les acteurs de secteur va malheureusement crescendo. Ils se sont engagés dans une partie de poker menteur et se renvoient la responsabilité de la guerre des prix, notamment dans les médias. Un coup d'oeil chez nos voisins suffit pourtant pour constater que les parties peuvent discuter et s'entendre sans recourir systématiquement à l'arbitrage du législateur. Loin de ces tensions et des pressions liées à la période de négociations commerciales en cours, j'espère que le Sénat saura construire avec sérénité et efficacité un cadre utile aux fournisseurs et aux distributeurs, dans l'intérêt de nos producteurs et des consommateurs. La commission des affaires économiques du Sénat a proposé trois évolutions majeures pour ce texte. Première nous avons choisi d'engager le débat sur l'usage du SRP+10, une manne financière versée depuis quatre ans aux distributeurs, dont l'efficacité en matière de redistribution aux agriculteurs n'a pas été démontrée par les rapports du Gouvernement et de l'inspection générale En effet, après quatre ans d'expérimentation, au cours desquelles ont régulièrement été dénoncées l'opacité et l'inefficacité du SRP+10 en matière de partage de la valeur, nous ne pouvions concevoir une reconduction de trois ans sans débat sur ce qui demeure une singularité française. Le texte issu de l'Assemblée nationale proposait de prolonger l'expérimentation jusqu'en 2026. En commission,

Pour résumer, le SRP+10 est aujourd'hui un chèque en blanc à la grande distribution, sans contrepartie garantie pour les producteurs. La commission a donc proposé de le suspendre pendant deux ans,

Cette position responsable de la part du législateur, qui doit s'assurer de la bonne application de la loi, témoigne aussi d'une exaspération, après quatre années sans transparence.

négocier plus durement pour conserver leur niveau de marge. Cette hypothèse est cependant à tempérer. Avec les dispositifs mis en place en 2022 par la loi Égalim 2, le contexte a changé. Je rappelle que la contractualisation écrite est devenue obligatoire et que les matières premières agricoles sont désormais non négociables : autant de dispositifs de protection traçables, vérifiables, qui ont fait leurs preuves, en conduisant dès 2022 à une revalorisation de 3,5 % de la rémunération des matières premières agricoles. Néanmoins, afin de tenir compte des préoccupations actuelles et de ne pas influer sur les négociations en cours, la commission propose de concilier les différents points de vue en acceptant la prolongation de l'expérimentation jusqu'en 2025,

Ce sont les fournisseurs qui financent ces promotions, rarement les distributeurs. Autrement dit, ils doivent vendre de plus en plus de volume à des prix de plus en plus cassés.

négliger ces milliers d'emplois et ces territoires dynamisés par la fabrication de ces produits, monsieur le ministre ? Après avoir fait tant d'efforts, notamment fiscaux, pour attirer des investissements étrangers, faut-il prendre le risque des délocalisations ? Autre inquiétude soulevée, l'encadrement des promotions sur les DPH pourrait avoir un impact sur l'inflation.

Le distributeur pourra donc, s'il le souhaite, augmenter le volume de promotion sur ces produits. L'encadrement que nous proposons vise principalement les 25 % qui font l'objet de surpromotions chocs.

tout en conservant le principe fondamental de liberté contractuelle. Nous pensons, en effet, qu'il n'appartient pas au législateur de se substituer aux parties et de dire à leur place quelle est la durée d'un préavis ou quel est le prix juste. Il ne nous appartient pas non plus de bouleverser structurellement le droit commercial en autorisant la rupture brutale des relations du La rédaction adoptée précise donc que, en cas d'échec des négociations au 1 mars, le préavis de rupture devra tenir compte des conditions économiques du marché, c'est-à-dire, par exemple, de l'inflation du coût des intrants ou du prix moyen accepté par les autres distributeurs concurrents. Ce faisant, nous répondons à une triple inquiétude : celle des PME, qui ne risquent plus d'être déréférencées subitement, puisque nous maintenons le principe du préavis ; celle des distributeurs, qui craignent de ne plus être livrés subitement ; celle des fournisseurs, qui ne sont plus obligés de livrer des produits à l'ancien tarif, c'est-à-dire à perte. Nous avons entendu les préoccupations de ceux qui estiment que le recours au juge pour faire appliquer la loi pourrait prendre trop de temps par rapport à la vie des affaires. C'est pourquoi la commission propose aujourd'hui une nouvelle rédaction tout en conservant les apports adoptés en commission. Nous avons ainsi un dispositif clair, souple, respectueux de la liberté des parties et tenant compte du contexte actuel.

depuis quinze ans, une guerre des prix s'est installée, fragilisant nos commerces et nos agriculteurs par la destruction de valeur. Je rappelle que cette loi,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation de l'agriculture française ne cesse de se dégrader Trop nombreux sont les agriculteurs qui ne parviennent pas à se payer décemment. Cette proposition de loi s'éloigne toutefois de notre coeur de cible issu de l'esprit des lois Égalim, à savoir garantir la juste rémunération des agriculteurs. Ce texte se concentre sur les relations entre les distributeurs et les fournisseurs. On peut donc légitimement s'interroger sur les conséquences pour les agriculteurs, qui sont en amont de la chaîne. de loi ne soit un énième essai, une nouvelle tentative face à l'inefficience des lois Égalim successives, en attendant une grande loi agricole censée, nous l'espérons, traiter les problématiques de fond. Pour l'heure, les dispositifs adoptés ces dernières années ont abouti à des échecs. Les auteurs de ce texte, issus de la majorité présidentielle, font le constat que la crise ukrainienne et la covid-19 ont rendu impossible l'atteinte des objectifs contenus dans les deux premières lois. Il faut l'admettre, ces événements n'ont pas aidé Mais la conjoncture n'est pas la seule responsable de ce manque de résultats. Le groupe socialiste avait alerté le Gouvernement sur le manque d'ambition de ces textes au vu de la gravité de la situation de notre agriculture. Notre priorité doit être de consolider notre modèle agricole, ainsi que les maillons qui constituent la chaîne de transformation et de distribution. Redevenir une véritable puissance agricole, assurer à nos concitoyens une alimentation française de qualité, garantir notre souveraineté alimentaire : ces objectifs, nous les approuvons sur de nombreuses Les atteindre n'est possible que grâce à un juste partage de la valeur. Agriculteurs, transformateurs, distributeurs, tous doivent trouver leur compte dans les négociations commerciales. Pour ce faire, notre rôle de législateurs est de veiller à une régulation et à une transparence totale de ces dernières. En cela, je salue l'article 1, qui vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit par la grande distribution, laquelle constitue des centrales d'achat à l'étranger pour ne pas être soumise aux règles encadrant les négociations commerciales telles que les ont fixées Comme l'a affirmé mon collègue député Gérard Leseul, notre rôle est de « corriger les dispositifs au fur et à mesure pour apporter un cadre qui permet de rééquilibrer ce qui est déséquilibré

nous considérons qu'une suppression pure et simple sans autre option n'est ni une solution opportune ni un bon signal donné aux acteurs de la négociation. Mes chers collègues, parce qu'elles sont, selon nous, un levier pertinent pour mieux rémunérer les agriculteurs dans les filières en difficulté, nous proposons de pérenniser les conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales qui lient une coopérative ou une organisation de producteurs, un un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Elles sont une alternative intéressante dans les filières peu allantes sur la contractualisation individuelle. Nous défendrons donc un amendement visant à revenir à la rédaction votée à l'Assemblée nationale, sur la proposition de nos collègues socialistes. En outre, nous proposons de rétablir le montant des taux de service mensuel pouvant donner lieu à des pénalités, mais à hauteur de 97 %. Mes chers collègues, la discussion de ce texte est l'occasion de remettre l'agriculture au coeur du débat public. Notre modèle agricole est en grande difficulté. La concurrence, l'absence de clauses miroirs, le manque d'attractivité du secteur sont d'autant de facteurs qui plombent notre agriculture. Pourtant, les enjeux auxquels nous faisons face nous imposent de trouver des solutions rapides et efficaces qui permettent à la France de se doter d'un modèle agricole efficient de loi n'est qu'une goutte d'eau. Elle doit s'inscrire dans une réflexion plus large, une réforme globale de notre modèle agricole. Je souhaite qu'un texte permette un rééquilibrage des relations entre industriels et distributeurs et qu'il ait, par ruissellement, des répercussions sur les producteurs. les producteurs. Après l'annonce par le Gouvernement d'une grande loi agricole dans les prochains mois, nous aurons, j'en suis convaincu, l'occasion de défendre la juste rémunération des agriculteurs.

Plusieurs facteurs expliquent cette inflation, à commencer par la situation internationale et les tensions qui la caractérisent : pandémie de covid-19, conséquences du réchauffement climatique sur les récoltes, agression de l'Ukraine par la Russie. Pour la production agricole, les crises de grande ampleur s'enchaînent et affectent toute la chaîne de valeur. Le coût des intrants et des matières premières s'envole, les tensions pour l'approvisionnement sont grandes. Du côté des entreprises agroalimentaires, la crise de l'énergie se répercute sur les coûts de production, dans un contexte où elles ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente. Pour les consommateurs et les consommatrices, qui sont au bout de la chaîne, c'est l'asphyxie : +60 % sur une bouteille d'huile, +22 % pour la farine, +20 % sur le paquet de pâtes, +16 % sur la volaille. La vie est chère, le caddie

Des produits plus chers, en moins grande quantité, ou tout simplement retirés du panier ... Cette situation ne peut plus durer, et pas plus pour les consommateurs et les consommatrices que pour les agriculteurs et les agricultrices. Mais il faut être honnête sur un point il y a des intérêts inconciliables. On ne peut pas, à la fois, faire baisser les prix pour les consommateurs, garantir des marges à la grande distribution, préserver des entreprises agroalimentaires intermédiaires, et assurer une juste rémunération aux producteurs et aux productrices. Aucun texte n'est capable de faire cela, parce que ce n'est pas possible L'intérêt des négociations commerciales- peu importe qui est autour de la table -, c'est d'avoir l'ascendant sur l'autre, de remporter l'avantage. Il n'y a pas de consensus possible entre la grande distribution, qui cherche à maintenir ses profits, et des entreprises intermédiaires qui doivent amortir leurs coûts. Il n'y a pas, dans ce système, de place pour le consommateur ou la consommatrice qui veut avoir accès à une alimentation de qualité à des prix raisonnables. Il n'y a pas non plus de juste rémunération du producteur et de la productrice, parce que la grande distribution n'est pas là pour ça. ça. On peut souhaiter travailler sur un seuil de revente à perte, mais il faut alors en faire un outil concret, et conditionner son existence à une obligation de résultat et de transparence des marges. Concrètement, il faut que ces 10 % fassent l'objet d'une évaluation, que l'on prouve qu'ils sont effectivement reversés aux producteurs et aux productrices. Si tel n'est pas le cas, si l'on établit que ces marges vont directement dans les poches de la grande distribution, alors ce mécanisme devra être supprimé.

Si nous avons l'objectif de mieux rémunérer nos agriculteurs et agricultrices, c'est une réforme en profondeur qu'il faut conduire. J'aborderai, en premier lieu, la politique commerciale. Quel est l'impact des traités de libre-échange sur nos producteurs et productrices ? J'entends souvent parler des exportations de la France prétendument permises par ces traités. Mais, concrètement, en termes de rémunération des filières françaises, sait-on mesurer la préférence du consommateur pour une viande moins chère venue de l'autre bout du monde ? Aucun bilan ne peut prouver que ces traités profitent aux producteurs et aux productrices ; pourtant, ils continuent d'être signés à tour de bras.

faisons des marchés publics le coeur d'une rémunération juste pour nos producteurs et productrices ; augmentons les seuils de la commande publique en circuits courts et en alimentation durable protégeons aussi nos agriculteurs et agricultrices des prédations de la grande distribution en imposant des prix planchers, avec un socle basé sur les coûts de production et un pourcentage en marge qui garantirait une rémunération minimale, quelle que soit la conjoncture.

sur des principes initiaux salvateurs. Je reviens rapidement sur certains d'entre eux. Égalim, c'est une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs du secteur, une plus juste rémunération de nos agriculteurs et, enfin, enfin, l'annonce de la fin des relations particulièrement conflictuelles entre acteurs de la distribution et fournisseurs lors de l'exercice redouté des négociations commerciales. La non-négociabilité des matières premières agricoles, le plafonnement des promotions sur les produits agricoles et l'encadrement de l'application des pénalités logistiques ont ainsi permis de façonner un dispositif robuste et prometteur, dans l'optique de rémunérer au juste prix La généralisation des contrats écrits et pluriannuels a permis d'opter pour une plus grande transparence en matière de négociation contractuelle et de construction des prix. Parallèlement, l'introduction dans les contrats d'une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l'évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l'énergie, a démontré toute sa pertinence. Malgré notre insistance, nous n'avions cependant pas été écoutés sur des sujets cruciaux. Nous avions tiré la sonnette d'alarme au sujet du phénomène d'évasion juridique et alerté à propos de l'encadrement déficient des marques de distributeurs. Le Gouvernement ne peut le nier aujourd'hui. C'est donc bien une loi Égalim 3 que nous examinons aujourd'hui, mes chers collègues. Il est en effet nécessaire de tirer les enseignements des dispositions législatives votées et de faire en sorte qu'elles s'appuient sur des fondations durables et pérennes. Le présent texte permet de mettre en lumière les défauts du droit en vigueur, tout en apportant les nécessaires éléments de réponse aux problématiques rencontrées par les acteurs sur le terrain. Ce sont des changements majeurs qui sont opérés, tant pour les consommateurs que pour les producteurs et les distributeurs. Les pratiques d'évasion juridique des grandes enseignes seront désormais plus durement sanctionnées. L'efficace plafonnement des promotions en valeur et volume a été prolongé et étendu aux aux produits de droguerie, parfumerie et hygiène. C'est un signal fort envoyé à l'ensemble de nos PME et de nos entreprises de taille intermédiaire (ETI). La période de renégociation contractuelle annuelle a été redessinée afin d'éviter toute asymétrie dans la relation commerciale. L'exclusion des fruits et légumes frais du dispositif SRP+10 était demandée par la profession ; nous l'avons prévue. Sur la disposition de majoration SRP+10, un débat s'est engagé, à juste titre, non pas sur la remise en question du dispositif final ni sur ses objectifs, mais sur son effet. Comme je l'ai précisé en amont, il est de notre devoir d'évaluer les dispositions législatives engagées pour mieux les conforter ou, si nécessaire, les adapter. Les producteurs ont-ils bénéficié de cette majoration ? La question mérite d'être posée. En tout cas, je le redis, il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir sur cette disposition. l'application des pénalités logistiques, cette arme ultime permettant à certains distributeurs mal intentionnés de réaliser des marges au détriment des producteurs, a été plus strictement encadrée et les sanctions en cas de pénalités frauduleuses ont été fortement durcies. de ce texte, le Sénat s'affirme plus que jamais comme la chambre de l'agriculture française et des agriculteurs. Cependant, je crois qu'il nous faut être prudents. Prudents, d'abord, face à la prolifération des normes, source d'une instabilité juridique pénalisant l'ensemble des acteurs du secteur. Prudents, ensuite, face à l'empilement de dispositifs juridiques qui peuvent manquer de cohérence et de lisibilité.

C'est en ayant à l'esprit cette exigence d'efficacité que la majorité des membres de mon groupe votera en faveur de la présente proposition de loi, car ce texte rétablit un juste équilibre entre fournisseurs et distributeurs. Nous voterons en faveur de cette proposition de loi, car elle pose les fondations d'une relation commerciale plus saine, à l'heure de l'inflation galopante ainsi que de l'envolée des prix des matières premières et de l'énergie, qui mettent à mal nos petites entreprises et nos agriculteurs. Nous voterons en faveur de cette proposition de loi, enfin, car elle permet de perfectionner le dispositif Égalim dans le cadre de notre volonté initiale

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

presque le même nombre de sénateurs dans l'hémicycle, nous entendons les mêmes orateurs exprimer les mêmes idées, les mêmes convictions. Pourtant, le contexte au fil des ans reste, lui aussi, le même : perte de compétitivité, perte d'exploitations, perte de foncier, perte de revenu. Nous ne pouvons que constater notre impuissance face à cette situation, face à cette érosion, et nous nous efforçons de poser un petit sparadrap au coup par coup là où cela fait le plus mal. Notre agriculture ne vaut-elle pas mieux ? Ne peut-on pas se poser pour réfléchir globalement ? La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été présentée dans les médias comme la loi Égalim 3. Je ne souscris absolument pas à cet intitulé ! Souvenez-vous, Égalim signifie « États généraux de l'agriculture et de l'alimentation ». On a perdu en route les États généraux : c'est bien dommage ! La méthode était la bonne : l'esprit initial était de mettre tout le monde autour d'une table, d'organiser une concertation avec tous les maillons de la chaîne pour qu'ils se parlent et prennent en considération la situation de chacun en vue du respect du coût de production, donc de l'agriculteur. Sous couvert du pouvoir d'achat des Français, on sait bien qui a supporté la charge de la guerre des prix : l'agriculteur et, au bout de la chaîne, le consommateur, car les produits d'appel ne sont que des leurres face aux marges réalisées avec les autres produits. Aujourd'hui que reste-t-il Un constat rappelé, dès le départ, par les auteurs de cette proposition de loi : « Pour la troisième fois en cinq ans, le législateur est amené à réglementer les relations entre fournisseurs et distributeurs, ce qui témoigne du climat de défiance qui règne lors des négociations commerciales. Il faut donc partir des enjeux et ensuite avoir une vision transversale pour les actions ; sinon, c'est de la stratégie à la petite semaine. Je déplore le manque de vision pour poser les enjeux : la souveraineté alimentaire, évidemment, mais aussi la santé que procure la qualité de notre alimentation, l'environnement, les emplois non délocalisables, le foncier, etc. Les problématiques sont transversales : comment assurer le bien-être de nos agriculteurs une agriculture raisonnée et rémunératrice ? Et comment, demain, donnerons-nous à manger aux 10 milliards d'habitants de la planète ? Nous devons être à la hauteur. Pour revaloriser ce métier, pour maintenir le nombre de paysans en France et- pourquoi pas ? -en gagner, il est urgent de définir une stratégie nationale avec les organisations professionnelles, l'ensemble des filières et tous les maillons de la chaîne. Les textes de loi se succèdent, mais ils sont rédigés dans un entre-soi. L'exemple du texte examiné aujourd'hui en est la preuve,

Certains veulent le maintenir, d'autres l'annuler ... L'incertitude sur ses effets positifs ou négatifs est telle que chacun y va de son analyse, sans véritable argument fondé. Les syndicats eux-mêmes ne sont pas en phase avec certaines filières. L'interprofession des fruits et légumes frais, Interfel, souhaite quitter ce dispositif alors que la Fédération nationale Si, comme la rapporteure l'affirme, les 600 millions d'euros qui devaient ruisseler vers l'agriculture ont été un véritable chèque en blanc offert à la grande distribution, pourquoi le syndicat majoritaire défendrait-il cette mesure ? C'est à n'y rien comprendre, et comment le législateur peut-il trancher sans l'avis de la profession ? Où est l'intérêt des agriculteurs ? Le texte que nous examinons resserre l'étau sur les distributeurs dans les négociations commerciales ; tant mieux. Mais si l'intention est louable, cela peut se retourner contre les agriculteurs français, car, demain, les quelques groupes qui se partagent la vente pourront faire le choix de produits étrangers moins chers.

Il y a donc urgence à reprendre un dialogue de raison et de conscience. Les distributeurs doivent comprendre les enjeux pour notre agriculture, mais aussi les enjeux d'image pour Face à des citoyens qui s'intéressent aux modes de production, aux étiquettes, nous pouvons coconstruire des modèles où chacun pourra tirer parti de la vente, ce que l'on appelle couramment un contrat « gagnant-gagnant ». Je l'ai dit la semaine dernière lors du débat sur la perte de compétitivité, nos voisins, que nous critiquons souvent, ont su mettre en place des organisations professionnelles collectives. Nos filières doivent s'unir pour ne pas être à la merci des distributeurs, car nos agriculteurs perdront toujours le combat entre une industrie agroalimentaire puissante, des organisations professionnelles trop nombreuses et une poignée de distributeurs qui sont toujours gagnants.

En 2020, déjà, j'évoquais les espoirs suscités par l'adoption d'Égalim, et les attentes déçues. Le groupe de suivi de cette loi, présidé par notre collègue Daniel Gremillet, a invité à en réviser le texte.

Aujourd'hui, nous sommes amenés, une nouvelle fois, à compléter ce texte. Notre objectif reste le même : garantir efficacement une juste répartition de la valeur et une juste rémunération de nos agriculteurs. Force est de constater, en effet, que le déséquilibre est exacerbé lors des négociations annuelles. Il est particulièrement accentué cette année par la crise énergétique et la pression inflationniste. La guerre des prix menée depuis de nombreuses années a contribué à la destruction de valeur

puisqu'il s'agissait de reconduire cette expérimentation. Nous devons nous assurer que le dispositif fonctionne correctement pour l'ensemble des maillons de la chaîne, de la production à la transformation et, bien évidemment, à la distribution.

et à y apporter des correctifs, notamment en demandant chaque année aux distributeurs un compte rendu détaillé,

Notre groupe a toujours défendu le partage de la valeur pour tendre vers une relation commerciale équilibrée, gagnant-gagnant. Avec la pression inflationniste actuelle, l'exercice n'est évidemment pas simple. Enfin, j'aimerais évoquer la question des pénalités logistiques. Celles-ci ont fait l'objet de riches débats en commission. Elles sont certes nécessaires pour garantir la réparation de certains préjudices, mais elles doivent être

pour exclure la filière des grossistes de l'application de ces règles, qui n'étaient pas adaptées à leurs spécificités. Malgré de textes successifs, les déséquilibres structurels demeurent forts, avec une distribution puissante et très concentrée. C'est pourquoi je pense qu'une vraie loi de régulation économique, apportant des correctifs à la loi de modernisation de l'économie, est toujours nécessaire. D'autres leviers doivent aussi être mobilisés pour soutenir notre agriculture et ses filières. Je pense notamment au projet de loi d'orientation et d'avenir de l'agriculture que vous préparez, monsieur le ministre,

chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour discuter de l'encadrement et de l'équité des relations commerciales dans le secteur alimentaire. Ce texte, qu'on appelle Égalim 3, montre qu'il est difficile de rééquilibrer les relations commerciales sans faire appel à des mesures structurantes. Dans un contexte de concurrence internationale, poussant au moins-disant social, environnemental et sanitaire, et de domination du marché par la grande distribution, les contournements et effets de bord des lois Égalim 1 et Égalim 2 sont nombreux. Et le secret des affaires rend plus complexe encore l'évaluation de l'efficacité ces textes. Il est plus que nécessaire de mettre en place des mesures structurantes pour rééquilibrer les rapports de force. Cela commence, nous le répétons, par le renoncement aux accords de libre-échange. La France doit aussi se battre activement pour la mise en place de clauses miroirs pour un meilleur contrôle des produits importés ne respectant pas nos normes. Nous sommes aussi convaincus qu'il est nécessaire de mettre en place au plus vite des mécanismes de régulation des marchés, et notamment des volumes au niveau européen. Alors que certaines enseignes semblent estimer que la pression sur les prix payés aux producteurs et fournisseurs est le moyen à privilégier pour garantir aux consommateurs un accès aux produits alimentaires, nous pensons au contraire qu'il convient de mener un travail structurel, je le répète, pour redonner leur valeur aux aux produits alimentaires et garantir un droit à l'alimentation, avec en perspective la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Un outil supplémentaire serait la rémunération des services écosystémiques rendus par les systèmes agricoles locaux et durables, qui permettrait d'améliorer le revenu des producteurs et rendrait plus accessibles à tous les produits de qualité. Enfin, Enfin, nous devons travailler à la relocalisation de l'alimentation par le soutien à la construction de filières locales et à la restauration collective. Tous ces éléments sortent du périmètre du texte que nous examinons aujourd'hui. aujourd'hui. Mais nous proposerons par amendement une mesure structurante, l'impossibilité pour un contrat entre agriculteur et acheteur de fixer un prix inférieur aux coûts de production, seule garantie pour un revenu paysan digne de ce nom. de ce nom. Si les solutions proposées par ce texte sont insuffisantes, nous considérons qu'elles permettent certaines avancées. Il est effectivement utile d'agir sur les pénalités logistiques, sur le contournement de la loi par des centrales d'achat à l'étranger, de tenter d'améliorer l'équité des relations entre fournisseurs et distributeurs et de viser à la sanctuarisation du coût des matières premières agricoles, en particulier pour les marques de distributeur. Sur le seuil de revente à perte, nous nous réjouissons qu'un compromis soit en vue, attendons beaucoup de l'évaluation de ses effets sur les marques de distributeurs. Il n'est pas normal que le ruissellement ne soit pas effectif. Même si nous ne croyons pas que ce texte apporte véritablement des solutions durables pour plus d'équité, notre vote sera favorable, en attendant de pouvoir véritablement travailler sur la réorientation

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons prétend apporter des réponses à l'industrie agroalimentaire contre les pratiques de la grande distribution, et plus particulièrement de la poignée de grands acheteurs qui se partagent actuellement le marché. En somme, nous assistons à un combat de géants contre des titans de l'alimentation- fournisseurs contre distributeurs -avec une concurrence féroce entre distributeurs, dont l'argument maître demeure l'accès aux prix les plus bas, et des fournisseurs qui se plaignent de l'explosion des coûts de l'énergie, des emballages, du transport, et de la matière première agricole. Ne soyons pas dupes, ce combat les conduit à bâtir leurs propres marges sur le dos des consommateurs et des agriculteurs : d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, tous ces intermédiaires font un maximum de profits L'organisation de pénuries de produits alimentaires dans un but spéculatif a pourtant bien été pointée, ici même, par notre commission des affaires économiques, qui a d'ailleurs réintroduit le mécanisme de relèvement du SRP pour éviter de replonger nos exploitants dans une nouvelle guerre des prix.

prétend faussement qu'il s'agit d'une loi Égalim 3, mais ceux qui sont en amont de la chaîne alimentaire ne ressentent toujours pas le « ruissellement » espéré. Dans un contexte chahuté par les aléas climatiques, la grippe aviaire, la guerre en Ukraine, la pénurie d'intrants et de matière de conditionnement, la production agricole française a certes progressé, selon l'Insee, de 17 % en valeur l'année dernière, mais, derrière

croule sous les chocs successifs, et demeure victime d'un rapport de force totalement inégal face aux mastodontes de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et le Gouvernement, qui soutient ce texte, d'annoncer, en même temps- enfin ! -une grande loi agricole pour le printemps ... La sécurité des approvisionnements de certains produits, qui manquent déjà dans les rayons des grandes surfaces, n'est pas près de se rétablir. Prenons garde, donc, à ce que cette loi ne permette pas aux industriels de l'agroalimentaire la répercussion de hausses qui pourraient avoisiner 20 %. Favoriser des hausses de prix pour gonfler la marge d'entreprises multinationales qui ne fabriquent pas en France, et qui iront verser des dividendes ailleurs, est inconcevable. Je doute que cette proposition de loi améliore notre souveraineté alimentaire, ni même qu'elle favorise la compétitivité de la ferme France. Alors que l'insécurité alimentaire gagne du terrain, que les ménages font face à une nouvelle poussée de l'inflation et, bientôt, à une nouvelle hausse des prix de l'énergie, que leur budget alimentaire est de plus en plus contraint, nous observons une descente en gamme dans le choix des produits. Nous espérions, à l'inverse, que vous exigeriez des grands industriels comme des distributeurs qu'ils compriment les hausses de prix et les amortissent afin de protéger le pouvoir d'achat des Français.

péril. Cessons de brader les intérêts des consommateurs ! La hausse des prix à laquelle ils feront face demain nous donnera, hélas ! raison, et n'aura d'autre intérêt que de faire la part belle à la malbouffe. La parole est

qui tue l'agriculture française. Il s'agit d'arrêter les surtranspositions, d'améliorer le cadre fiscal pour favoriser l'investissement et d'encourager l'innovation au service de la productivité, pour faire qu'enfin les agriculteurs aient confiance et qu'enfin les Français soient fiers de leur agriculture, la dessinent, le disent

le prix défini ne puisse être inférieur au coût de production. Il n'est pas acceptable en effet qu'un agriculteur puisse vendre en dessous de son prix de revient. C'est pourtant ce qui continue de se passer pour bon nombre de producteurs, malgré l'obligation de prise en compte des indicateurs des coûts de production dans les contrats prévus par la loi. Ainsi, la filière bio connaît des difficultés économiques

C'est la preuve qu'Égalim 2 n'a pas porté ses fruits. Certes, cette mesure est complexe à mettre en oeuvre, car le coût de production varie, mais la définition des indicateurs prévus par la loi Égalim 2 devrait permettre de fixer ce prix de revient, tout en respectant la liberté contractuelle des deux parties et en s'adaptant à la diversité des situations et des filières. Il s'agit d'affirmer un principe fort : permettre un revenu minimal agricole, en s'assurant qu'un contrat ne puisse imposer à un agriculteur de vendre à perte.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à préciser la définition du coût de production pris en compte dans les contrats prévus par la loi Égalim 2. À défaut d'une interdiction de conclure un contrat rémunérant l'agriculteur au minimum au prix de revient, il convient de s'assurer que le coût de production pris en considération dans les contrats tienne compte d'une rémunération équitable de la main-d'oeuvre agricole, salariée et non salariée. Comme nous l'avons souligné, aujourd'hui encore, de nombreux contrats sont conclus sans garantir une couverture de l'ensemble des coûts de production, en particulier les coûts de main-d'oeuvre. Dans ce contexte, préciser la définition du coût de production semble utile, pour pousser à une contractualisation plus juste, permettant aux producteurs de vivre dignement. Quel

Vous parlez de pertinence. Dans tous les domaines, le coût salarial doit forcément être pris en compte, puisqu'il constitue la base du coût de production. Notre

Il aurait été pour moi inconcevable, comme cela a été un temps envisagé, de suspendre un mécanisme demandé par les agriculteurs, et ce au nom de la lutte contre l'inflation. Chacun sait qu'il nous faut lutter contre la vie chère, qui pénalise nos concitoyens, mais l'idée que cette lutte se fasse au détriment de la rémunération des agriculteurs m'est extrêmement désagréable. L'image que nous avons donnée lors de l'examen du texte me semble dommageable pour notre assemblée. D'une certaine manière, nous avons pu donner l'impression que négocier les fins de mois des agriculteurs pour gagner quelques dixièmes de points d'inflation était une idée moralement acceptable. Je ne peux m'y résoudre. Il n'est pas imaginable de troquer le fruit du travail effectué par nos agriculteurs pour la poursuite d'un objectif de réduction des prix qui, nous le savons, ne sera pas rempli par la suppression du dispositif SRP+10. Dans l'un de ses rapports, l'inspection générale des finances chiffre l'impact du mécanisme SRP+10 à 0,17 % d'inflation, soit une infime partie de la hausse des prix constatée dans les rayons aujourd'hui. Ce n'est pas rendre honneur au labeur des agriculteurs que d'avoir proposé une telle suspension du SRP+10. La valeur travail, que le Sénat a toujours défendue, doit rester pour nous un véritable totem. Ainsi, vous l'aurez compris, mes chers collègues, je suis ravi que notre rapporteure ait accepté de rejoindre les positions exprimées par la quasi-intégralité des groupes politiques visant à maintenir ce dispositif essentiel pour les agriculteurs. Cette issue

Par cet amendement d'appel, nous voulons relayer les craintes de nombreux syndicats agricoles de voir le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte simplement suspendu, sans préavis, alors même que les négociations commerciales en cours sont particulièrement virulentes. Ils refusent d'être de nouveau une simple variable d'ajustement dans la guerre des prix que se livrent fournisseurs et distributeurs. Comme le rappellent la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, nous ne pouvons pas affirmer que le SRP est la cause de l'inflation actuelle des prix alimentaires. Ce mécanisme apporte de l'oxygène aux négociations commerciales ; il constitue un barrage à la guerre des prix entre distributeurs et nous permet d'éviter de retomber dans la spirale de baisse du revenu des producteurs.

Nous avons toujours été constants- je l'ai dit -dans nos positions concernant ces lois. Nous estimons qu'elles ne vont pas assez loin, qu'elles ne sont pas assez coercitives et qu'à vouloir ménager toutes les parties nous ne donnons pas un cadre réellement protecteur aux agriculteurs qui sont ceux qui souffrent le plus de la guerre des prix. Le SRP+10 n'aura pas atteint les objectifs initiaux pour lesquels il a été institué, à savoir une meilleure rémunération des agriculteurs. Nous considérons que le ruissellement tant tant attendu n'est pas au rendez-vous et que les premières victimes se situent toujours en amont de la chaîne. En conséquence, si nous estimons que le maintien du dispositif à court terme est la moins mauvaise des solutions, il nous semble dans le même temps évident qu'il faudra procéder très rapidement à une nouvelle remise à plat des lois Égalim. La parole est à M.

Cet amendement de repli vise à rétablir le dispositif SRP+10 pour une période de deux ans et à prévoir une évaluation annuelle permettant de tirer les conclusions définitives de sa mise en oeuvre. Il reprend ainsi les dispositions de l'article 2 supprimé en commission, qui prévoyait la remise chaque année d'un rapport d'évaluation. Par ailleurs, il tend à exclure les fruits et légumes frais de l'application du SRP+10, tout en permettant au ministre, par arrêté, de réintégrer certains de ces produits dans le champ d'application de la mesure.

... En l'absence de résultats probants en termes de meilleure répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire, nous estimons qu'à terme il faudra nécessairement réformer ce dispositif. D'où notre proposition de maintenir le SRP+10 pour une période de seulement deux ans.

Est-ce qu'il est à l'origine d'une hausse des prix qui ne profite qu'aux distributeurs et industriels les plus puissants ? Pour certains, cette disposition considérée comme un cadeau à la grande distribution a entraîné une inflation estimée en 2019 à 1,6 milliard d'euros sur deux ans- c'est la position des associations de défense de consommateurs, en particulier l'UFC-Que Choisir. Pour d'autres, en revanche, sa remise en cause à la veille de la clôture des négociations commerciales entraînerait de nouveau une guerre des prix préjudiciable aux agriculteurs. La vérité, c'est que nous n'avons pas d'études fiables pour évaluer les impacts de ce dispositif sur les dernières années. C'est pourquoi nous proposons, à l'instar de Mme Loisier, de prolonger l'expérimentation du SRP+10 jusqu'en 2025, en excluant les fruits et légumes et en imposant une évaluation fine de l'impact de ce dispositif. Nous ne pensons pas que ce mécanisme pourra régler la question du partage de la valeur entre les acteurs de l'agroalimentaire. Il reste une rustine, le déséquilibre étant structurel du fait de la configuration même du secteur agroalimentaire. Comment pourrait-il en être autrement, alors que d'un bout à l'autre de la chaîne nous avons les agriculteurs, nombreux, mais peu organisés pour négocier, quelques groupes de distribution regroupés en centrales d'achat très puissantes et, entre les deux, des acteurs industriels de taille intermédiaire qui subissent de surcroît la hausse des prix de l'énergie Il n'empêche qu'il faut protéger la partie la plus fragile de ce système de négociations commerciales libéralisé : les agriculteurs. C'est le sens de notre amendement de compromis et d'équilibre. La

de l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

pour soutenir l'amendement n° 38. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas : ne pas vouloir supprimer le SRP+10 sur les fruits et légumes est une aberration Annuellement, cela coûte 30 millions d'euros à la filière tomates, 25 millions d'euros à la filière pommes-poires, 6 millions d'euros à la filière carottes, 4 millions d'euros à la filière asperges, 11 millions d'euros à la filière melons, 15 millions d'euros à la filière fraises. Soit 91 millions d'euros perdus chaque année, et cela depuis quatre

le principe de non-discrimination tarifaire, actuellement applicable aux seuls produits agricoles et agroalimentaires, à l'ensemble des produits de grande consommation. L'objet du principe de non-discrimination pour les produits agroalimentaires est de renforcer le tarif du fournisseur en précisant le contenu des conditions particulières de vente justifiant les services de coopération commerciale rendus par le distributeur. Ce dispositif est justifié par le contexte concurrentiel spécifique du secteur agroalimentaire. Il ne me semble pas justifié d'étendre à tous les secteurs du commerce des dispositions spécifiques à la filière agroalimentaire. Par ailleurs,

de « surmarges » réalisées par les grandes surfaces. Dans un contexte d'inflation et de turbulences pour la filière biologique, la FNSEA elle-même a dénoncé ces pratiques

d'aller plus loin encore, en étudiant la possibilité d'un encadrement de ces « surmarges ». Il s'agit de ramener de la justice dans l'accès aux produits de qualité et de connaître le réel ordre de grandeur de la différence de coût entre produits conventionnels et produits sous Siqo,

peu paradoxal : si certaines PME n'avaient que les promotions pour rivaliser avec les grandes marques connues du grand public, ce n'est pas tant l'encadrement des promotions en volume qu'elles devraient chercher à supprimer

Ainsi, certains syndicats représentant des PME estiment que, à l'instar d'autres dispositions des lois Égalim 1 et 2, l'encadrement des promotions en volume peut avoir des effets contrastés pour certaines petites entreprises et les défavoriser par rapport aux grands groupes. doit donc permettre de caractériser ces problématiques et de proposer des adaptations de ces mesures qui permettent à la fois de protéger le revenu des agriculteurs et de garantir une concurrence loyale entre les entreprises, quelle que soit leur taille. Cet amendement vise également à obtenir, ce rapport, des informations sur les effets de l'encadrement des promotions sur le revenu agricole et la répartition des marges, cet impact restant à ce jour encore difficile à caractériser. Il est important d'encourager une plus grande transparence pour favoriser le fameux

le texte sur l'initiative de nos collègues députés socialistes, mais malheureusement supprimée en commission par Mme la rapporteure, qui lui a préféré le maintien de leur expérimentation jusqu'au 31 décembre 2025.

Cette analyse ressort également du rapport d'information sur l'évaluation de la loi Égalim publié le 23 février 2022 par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui préconisait la pérennisation Nous regrettons donc le choix de notre rapporteure, qui n'a pas voulu envoyer un signal positif en faveur de la généralisation, quand cela est possible et nécessaire, de ce type de convention.

commission ? Nous sommes d'accord quant à l'intérêt de ces conventions tripartites. Simplement, leur pérennisation nous semble trop précoce à l'heure qu'il est, puisque nous n'avons aucune évaluation véritable de ces conventions et que nous ne savons pas si les soucis de concurrence

reviendrait à supprimer le principe même de négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur, puisque l'on rendrait illégal le fait pour un distributeur de ne pas accepter tout simplement le tarif proposé par le fournisseur. Un débat similaire a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous cherchons plutôt à rééquilibrer les relations entre distributeurs et fournisseurs. Le risque est là de passer d'un extrême à l'autre.

S'il n'y a pas d'accord à cette date, c'est le préavis de rupture qui prend le relais, préavis durant lequel les fournisseurs doivent continuer de livrer à l'ancien tarif. La version initiale de la proposition de loi, soumise à l'Assemblée nationale, précisait que ce serait Canévet par l'amendement n° 3 rectifié , le tarif demandé par le fournisseur qui s'appliquerait durant ce préavis. En séance, les députés sont revenus sur ces dispositions et ont décidé qu'en l'absence d'accord au 1 mars, il y aurait rupture brutale des relations, c'est-à-dire arrêt immédiat des livraisons.

très peu d'acteurs et de négociations commerciales : c'est l'épaisseur du trait, à savoir les rares entreprises qui n'auraient pas conclu d'accord au 1 mars, qui n'en auraient toujours pas trouvé à l'issue d'une médiation et qui auraient face à elles un distributeur qui, visiblement, ne respecte pas la loi.

s'il y a toujours désaccord et si les parties saisissent le juge, celui-ci devra lui-même statuer selon la procédure accélérée au fond : il prendra une décision rapide- nous l'espérons,

contraignant ainsi le choix des parties. Enfin, si je comprends bien, vous souhaitez que les conditions du préavis de rupture soient déterminées en tenant compte de la situation économique. Dans ce cadre, la prise en compte, dans la médiation, du prix convenu entre le fournisseur et d'autres

le médiateur des relations commerciales agricoles, avec lequel nous avons travaillé et réfléchi à ces dispositions. Je pense que nous pouvons continuer cette réflexion avec vous, avec les députés et avec le médiateur, pour trouver le Graal

Les sénateurs du groupe socialiste estiment en effet que la situation sanitaire, économique et géopolitique que nous connaissons depuis 2020 engendre de forts dysfonctionnements dans la chaîne d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Or de nombreux acteurs de la chaîne demandent le maintien de ces taux dans la loi, mais à des niveaux revus à la baisse. Nous considérons que, sur ce sujet, il faut faire preuve de précaution et mener des évaluations.

taux de service. Cela dépend d'énormément de facteurs- la situation internationale, le type de produits, la taille du fournisseur, la période de l'année, etc. Il est impossible de trouver un taux unique qui soit juste pour les dizaines de milliers de références qu'on trouve dans un supermarché.

le ministre. Cet amendement vise à réintroduire le mécanisme voté par l'Assemblée nationale permettant au Gouvernement de suspendre, en cas de crise d'une ampleur exceptionnelle, l'application des pénalités logistiques. Il ne vous a pas échappé qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir anodin, compte tenu de l'ampleur nationale de la suspension des pénalités logistiques. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder par décret en Conseil d'État, dont la consultation me semble indispensable pour veiller à la stricte proportionnalité d'un tel dispositif.

pour certains secteurs. Autrement dit, vous ne l'autorisez qu'à l'échelle globale et vous supprimez la possibilité de renouveler la période de suspension. La commission émet donc un avis défavorable

18 est présenté par le Gouvernement.

que ces dernières n'ont pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles. Si l'intervention du tiers indépendant est une innovation intéressante, qui facilite les négociations commerciales,

et le sous-amendement

Il nous semble néanmoins que, depuis les négociations commerciales de 2021, un certain nombre d'éléments ont été apportés, d'abord lors de l'examen de la loi Égalim 2, qui a renforcé l'encadrement des contrats. Depuis les négociations de 2021-2022, les contrats portant sur les MDD doivent intégrer une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole. D'autres mesures sont désormais obligatoires, comme l'engagement du distributeur sur un volume prévisionnel de production et la définition d'une durée minimale de préavis. En outre, il est désormais interdit pour un distributeur

qu'est passible d'une amende le fait « pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur, sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier

de la mise en place d'un mécanisme d'évaluation fine des véritables bénéficiaires du relèvement du seuil de revente à perte ou de la réécriture de l'article 3, qui permet de ne pas laisser les fournisseurs sans solution en cas d'échec des négociations

d'accroître l'accessibilité à une alimentation saine et durable ou de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Malheureusement, l'adoption de cette proposition de loi ne suffira pas à endiguer les hausses consécutives à l'envolée prix des matières premières agricoles et industrielles ni à éviter la disparition d'entreprises, les destructions d'emplois et les ruptures de production. Nous avons besoin non pas d'une énième loi technocratique, mais d'un changement de méthode. Or nous en sommes loin. La

loyales, sans opter pour le moins-disant environnemental et social. Le panier alimentaire ne doit pas être la variable d'ajustement dans un budget serré. La solution est de redonner du pouvoir d'achat aux plus défavorisés. Il faut arrêter avec le bas de gamme pour les moins favorisés, qui provoque obésité, diabète et leurs corollaires de maladies graves. Cette proposition de loi est un petit pas vers un meilleur partage de la valeur, vers une évaluation de cette répartition. C'est un petit pas : clairement, nous travaillons à la marge, dans tous les sens du terme.

monsieur le ministre, mes chers collègues, loin du vacarme médiatique et des pressions en tout genre, nous avons ce soir achevé l'examen d'une proposition de loi qui Si la presse lui a parfois attribué le nom d'« Égalim 3 », c'est bien parce que les deux premières lois éponymes n'avaient pas complètement atteint leurs objectifs initiaux. Je ne sais pas si le texte dont nous venons de discuter y parviendra davantage je sais en revanche que les dispositifs votés au Sénat, fruits du travail du groupe de suivi d'Égalim, permettront de faciliter quelque peu les relations commerciales, que nous savons tendues, particulièrement en cette période d'inflation.

Je salue également le travail d'orfèvre de la rapporteure, qui nous a proposé à l'article 3 un système innovant pour régler les cas où les négociations commerciales annuelles échoueraient au 1mars. Il laisse une plus grande place à la médiation et prend en compte les conditions de marché pour toute signature de préavis. Enfin, les amendements adoptés sur l'initiative de nos collègues Daniel Gremillet et Laurent Duplomb sur la non-négociabilité des matières premières agricoles pour les produits vendus sous marques de distributeurs sont une avancée capitale. Ils parachèvent ainsi la sanctuarisation, entamée dans la loi Égalim 2, du prix des produits de nos agriculteurs. D'autres avancées sont à saluer, notamment l'encadrement des pénalités logistiques et le durcissement de notre législation à l'égard des centrales d'achat européennes. Le Sénat a une nouvelle fois apporté sa pierre à l'édifice et complété un texte qui était lacunaire lors de son dépôt à l'Assemblée nationale. À la veille du salon de l'agriculture, nous envoyons par ailleurs un signal fort de soutien à tous nos agriculteurs, pour que le fruit de leur travail soit rémunéré En conclusion, le groupe Les Républicains votera ce texte, qui est attendu par de très nombreux acteurs. La

Cette question, ainsi que celle de la diversité des modèles agricoles français, de leur complémentarité, de leur compétitivité,

vers l'agroécologie. Je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens, tout en répondant aux enjeux de compétitivité qui se posent de manière accrue et problématique à l'ensemble de la ferme France. Il faudra composer

Merci,